fera une déclaration, en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre, suivie d'un débat et d'un vote, demain à Acte est donné de cette demande. En conséquence, le Gouvernement demande que le Sénat siège ce vendredi 2 avril, matin, après-midi et soir pour poursuivre l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 7 avril après-midi, après les questions d'actualité au Gouvernement, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés. Acte est donné de ces demandes. Nous pourrions prévoir pour ce texte une discussion générale de 45 minutes.

L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

permettez-moi tout d'abord de vous dire qu'il n'y a pas de tri, et que ce mot devrait être banni de notre vocabulaire à ce stade de la crise. Dites-le aux familles de que nous traversons nous mobilise maintenant depuis un an et demi, en France comme ailleurs. Nous avons eu à développer des réponses mesurées et évolutives face à la situation que nous connaissons, mais nous avons aussi un devoir de transparence vis-à-vis des Français.

La réalité, c'est aussi que la situation sanitaire demeure plus que préoccupante : plus de 29 000 Français sont hospitalisés en raison du covid et les patients atteints du virus occupent 89 % des lits de réanimation,

Cette action, vous la connaissez, elle s'appuie sur la gestion quotidienne de l'ensemble des ressources dont nous disposons au regard de l'évolution de la situation sanitaire. Concrètement, elle permet de déployer des outils- masques, gels, vaccins -dont nous avons besoin, assurer que ceux-ci aillent où il faut, quand il le faut, grâce à une logistique d'ampleur. Notre réponse est territorialisée, concertée, en fonction de la situation vécue dans chaque région. Nous rendons compte en toute transparence, en temps réel, chaque semaine, nous échangeons dans cet hémicycle quand la situation l'exige, M. le Président de la République s'adresse à nos concitoyens, ce qu'il entend faire ce soir. Vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas de préjuger de ses propos néanmoins, en complément des temps dédiés, le Premier ministre a fait le choix d'ouvrir un débat parlementaire dès demain pour que nous puissions échanger plus largement, en toute transparence, sur la réponse la plus adaptée à la situation que nous connaissons. Monsieur le sénateur, les Français attendent mieux que de vaines polémiques. Hissons-nous à la hauteur de l'enjeu pour sortir collectivement plus forts de cette crise. Madame la ministre, vous pouvez bannir un mot du vocabulaire, mais vous ne le bannirez pas de la réalité ! En déprogrammant plus de 80 % des interventions dans les hôpitaux,

La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, nous savons que la troisième vague est très grave et nous sommes une nouvelle fois, en élus responsables, aux côtés de tous nos soignants, soucieux de continuer à appliquer les gestes barrières. Pourtant, la situation sanitaire n'interdit pas d'envisager l'avenir, même proche, non plus que de faire des projets collectifs, comme les prochaines élections. Depuis plus d'un an, les élus et les candidats aux élections départementales et régionales vont, comme Ulysse, de report en report, de faux départ en faux espoirs. Ils ne sont pas, à ce titre, pleinement mobilisables sur la durée pour appuyer les plans de relance et pour être aux côtés de celles et de ceux qui vivent la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Les exécutifs attendent. Lundi, le conseil scientifique, comme la loi du 23 février 2021 le prévoit, a émis un avis concernant un possible nouveau report des élections départementales et régionales, dont nous venons pourtant d'adopter le report en juin. Les élus, mes chers collègues, ressentent encore l'amertume des conditions de préparation si incertaines des élections municipales de mars 2020. Nous ne pourrons pas forcément réitérer un tel exploit. Comme n'hésitait pas à le dire François Mitterrand, l'action politique à certaines heures est comme le scalpel du chirurgien : elle ne laisse pas de place à l'incertitude. Aussi, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de nous proposer très vite une date fixe, un projet de loi, un calendrier, un débat parlementaire, ainsi qu'une promulgation rapide. Nous souhaitons sacraliser le moment de la campagne électorale et de la confrontation des projets, qui est, mes tout en assurant la sécurisation sanitaire et juridique des candidats, électeurs et personnels. Pour le moment, une campagne électorale sans contact, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Nous vous demandons également de prévoir dès à présent des conditions permettant de nous adapter à toutes les situations de crise. Mes chers collègues, les élus départementaux et régionaux sont indispensables pour affronter ensemble et rapidement les moments très difficiles qui s'annoncent. Monsieur le Premier ministre, dedans avec les miens, certes, mais serons-nous en juin citoyens

est à Mme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, le conseil scientifique, vous l'avez rappelé, a reçu mandat d'émettre un avis sur le déroulement du scrutin démocratique en période d'épidémie. Il a mené un travail difficile et remarquable que je veux ici saluer, malgré les différentes incertitudes

pour notre démocratie. Après un an de crise sanitaire, nous comprenons la lassitude et, parfois, l'incompréhension des Français à l'égard de ces questions. La responsabilité du Gouvernement est de prendre des décisions souvent difficiles, mais toujours nécessaires pour la santé des Français. Le report ou le maintien des élections est une décision lourde de conséquences. Le Premier ministre, Jean Castex, va lancer des consultations afin d'aboutir à une solution compatible avec la protection de chacun contre l'épidémie, mais aussi avec les impératifs démocratiques. Pour cela, nous rechercherons le consensus politique le plus large possible avec l'ensemble des partis et des groupes représentés.

dernier, le fabricant de silicium Ferropem annonçait la suppression de 360 emplois en Savoie et en Isère. C'est un savoir-faire centenaire qui est menacé. Le silicium est un produit essentiel pour de nombreuses activités industrielles, notamment pour la fabrication de panneaux photovoltaïques. En Isère toujours, c'est l'entreprise Photowatt, l'un des rares producteurs français de panneaux solaires, ses 215 salariés et leur immense savoir-faire, qui sont également menacés. Après avoir acheté ses panneaux solaires en Chine pendant des années, sa maison mère, EDF, se désengage. On marche sur la tête ! Sur l'autel de la rentabilité capitaliste, c'est toute la filière photovoltaïque française, voire européenne, qui est sacrifiée. L'énergie solaire est pourtant indispensable, tant pour la transition énergétique que pour la souveraineté de la France. Ne plus produire de panneaux photovoltaïques en France, c'est aggraver notre bilan carbone et notre dépendance à la Chine. Un comble en pleine discussion Cela témoigne de l'absence totale de stratégie en matière de transition énergétique de la France. L'ombre colossale d'Hercule plane sur cette triste affaire. Alors que l'on s'apprête à nationaliser et à financer à fonds perdu la filière nucléaire, qui ne sera jamais rentable, on continue à confier au privé tout l'effort de transition énergétique. Sacrée réussite : nous sommes déjà en retard sur les objectifs 2020 ! Monsieur le Premier ministre, allez-vous agir pour sauver le panneau solaire français ? Allez-vous enfin déployer une stratégie publique de développement des énergies renouvelables et respecter les objectifs de votre Allez-vous consulter le Parlement et le peuple avant d'engager, avec le projet Hercule, l'avenir énergétique de la France pour les trente prochaines années ?

sujet majeur : la production d'électricité photovoltaïque et ses conséquences industrielles pour notre pays et pour l'Europe. Vous l'avez rappelé, nous avons des ambitions fortes,

question renvoie à un autre sujet, celui de l'origine des panneaux, des tuiles et des cellules photovoltaïques

Nous devons changer cela. Vous vous souvenez que, pour encourager la consommation d'électricité d'origine photovoltaïque, plusieurs gouvernements successifs avaient augmenté les tarifs d'achat,

qui a longtemps manqué, nous la mettons progressivement en place. D'abord, nous veillons à ce que tous les appels d'offres pour l'achat de ces matériels comportent des critères en matière de contenu carbone, afin de favoriser les panneaux les plus performants, c'est-à-dire produits avec l'impact climatique le plus réduit, ce qui conduira, vous le savez, à écarter un certain nombre de ces produits importés qui ne répondent pas à ses conditions. Ensuite, cette stratégie industrielle doit aussi être menée dans un cadre européen et nous travaillons avec la Commission sur la possibilité d'introduire des critères de contenu de production locale dans tous

pour le lancement d'une alliance européenne pour le photovoltaïque, qui entre exactement dans les objectifs que vous avez appelés de vos voeux, alliance européenne qui a été annoncée par la ministre déléguée chargée de l'industrie le 22 février dernier, aux côtés du commissaire chargé de l'énergie.

que nous avons sauvé. Lorsque j'ai pris mes fonctions de chef du Gouvernement, vous avez raison de le rappeler, EDF voulait fermer Photowatt, nous l'en avons empêché,

mesdames, messieurs les sénateurs, ce gouvernement est pleinement mobilisé pour la construction d'une filière photovoltaïque souveraine et durable.

La version 2021 est marquée par la réforme de la fiscalité locale avec, d'une part, la fin de l'encaissement de la taxe d'habitation par les communes et, d'autre part, le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière

est égal à 1 plus la ressource à compenser moins la ressource de compensation divisée par la taxe foncière sur les propriétés bâties après réforme ». Je m'arrête là. Ce document est un véritable chef-d'oeuvre de l'administration fiscale, aussi compliqué à comprendre qu'une attestation dérogatoire. Vous le savez, cette réforme suscite chez de nombreux élus des inquiétudes sur la compensation de la taxe d'habitation. C'est pourquoi un effort de clarification est nécessaire sur la détermination du coefficient correcteur. Monsieur le ministre délégué, le Gouvernement doit prévoir un exercice de simplification et d'explication à destination des maires. J'ajoute que, en fin d'année, les Français vont recevoir leur feuille d'impôts locaux de laquelle, pour 80 % d'entre eux, la taxe d'habitation disparaîtra. Il restera le foncier bâti, qui figurera sur une seule ligne avec un seul taux, résultant de l'addition du taux communal et du taux départemental. Les maires, comme toujours, seront directement responsables devant les habitants. Par souci de transparence, il est indispensable qu'une clarification soit faite auprès du contribuable afin que celui-ci n'ait pas l'impression que la commune a augmenté massivement son taux d'impôt foncier en contrepartie de la suppression de la taxe d'habitation décidée par l'État. Merci, monsieur le ministre, de nous apporter des précisions en la matière.

quelques mots pour répondre à votre question et, d'abord, pour vous rassurer : l'état 1259 n'a pas fondamentalement changé par rapport à l'année dernière et porte toujours, pour les communes, les informations les plus précises possible sur les recettes prévisionnelles en matière de fiscalité, afin de leur permettre de bâtir leur budget.

Quelle est la principale différence ? Elle tient à la mise en oeuvre de la réforme de la taxe d'habitation. Cela passe par deux canaux, dont le calcul du coefficient correcteur, dont vous avez rappelé la formule telle qu'elle est littéralement expliquée. Il s'agit, en réalité, d'une règle de trois : lorsque les ressources attribuées depuis le département sont égales à 100 et que la ressource précédente de la collectivité

auprès de chaque maire pour expliquer les différences. Concernant la taxe foncière, il y a effectivement addition des taux, comme nous l'avions annoncé, mais le montant total de la taxe foncière sur les propriétés bâties reste strictement le même, nonobstant d'éventuelles évolutions de taux décidées par telle ou telle des collectivités désormais attributaires de cette taxe. À taux constant, le montant payé par le contribuable

les 20 % de ménages continuant à la payer bénéficieront d'une première baisse d'un tiers. Il y a toujours deux feuilles d'imposition locale : une pour feu la taxe d'habitation et une pour la taxe foncière. Il n'y aura donc pas de confusion. Je le répète, l'ensemble des maires recevront une explication plus détaillée, peut-être plus littéraire, de l'état 1259, qu'ils ont reçu récemment. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. « Je viens d'avoir 32 ans et je me suis fait vacciner. La logique aurait voulu que mes parents le soient avant moi, mais ils n'ont pas la chance de vivre aux États-Unis. » Tels sont les messages que nous recevons. ainsi, monsieur le Premier ministre, qu'est vue la France, cinquième puissance mondiale. Depuis un an, nous vivons au rythme des confinements et des déconfinements, de la fermeture des écoles et des commerces et du triste décompte des entrées en réanimation et des morts. Un an plus tard, nous avons le sentiment que rien n'a changé, que rien n'a évolué et que, malgré votre assurance et volonté de tout faire seuls, sans concertation, vous n'avez tiré aucun enseignement de vos erreurs. L'année dernière, vous nous promettiez 14 500 lits de réanimation. La vérité est qu'il n'y en a que 6 733. L'association entre le public et le privé ne se fait toujours pas. Un an plus tard, la solution vaccinale existe, mais, en France, seulement 3,9 % population est vaccinée contre 50 % aux États-Unis, 60 % en Grande-Bretagne, et même 85 % en Israël. Si nous nous comparons à d'autres pays, ce que vous aimez faire quand cela vous est flatteur, nous voyons donc que nous pouvons mieux faire. pouvons mieux faire. Monsieur le Premier ministre, pendant combien de temps allez-vous nous faire vivre au rythme de ces annonces toujours plus pessimistes les unes que les autres ?

nous adapter, évaluer et faire évoluer les protocoles, les doctrines, parfois en poussant les murs, parfois en transformant les industries pour créer des masques, du gel hydroalcoolique, maintenant des vaccins, avec une logistique considérable. Il nous a fallu agir avec méthode et avec transparence, qui nous a permis d'obtenir des résultats que nul ne croyait possibles il y a encore quelques semaines. Concrètement, plus de 8,2 millions de personnes ont bénéficié d'au moins une injection et 2,8 millions de deux. Peut-être pourrions-nous nous féliciter ensemble

collectif dont nous devrions nous réjouir et qui nous place en tête des pays européens sur la vaccination des personnes les plus âgées. C'est un tour de force, rendu possible par la mobilisation de tous les acteurs et par l'accélération de notre campagne vaccinale.

en priorisant les publics les plus fragiles et les plus exposés, en démultipliant les canaux avec l'ouverture de mégacentres dédiés, avec le concours des forces armées, en montant en puissance avec les centres de vaccination existants sur les territoires, ... Il faut conclure. ... en mobilisant tous les professionnels de santé possible et en allant vers les

La vérité est donc là ! Notre problème, monsieur le Premier ministre, est que la France est gérée par la peur et la division parce que vous avez vous-même peur de prendre des risques. que vous avez attendu de voir le résultat des campagnes de vaccination dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne pour juger des effets secondaires et pour, enfin, commander les vaccins et organiser leur administration. Aujourd'hui, vous nous annoncez que vous allez mettre en place des « vaccinodromes », alors que nos professionnels de santé ont mené une campagne de vaccination contre la grippe de façon remarquable. C'est ce Les Français sont fatigués des effets d'annonce et attendent aujourd'hui des actes. Gouverner un pays, c'est fédérer ses habitants pour lutter et combattre. Ayez la modestie de reconnaître vos erreurs comme l'a fait Angela Merkel,

En tant que président du groupe d'amitié France-Afghanistan, il est de mon devoir d'exprimer notre inquiétude concernant la situation dans ce pays. Le retrait des troupes américaines, prévu au 1 mai, fait craindre une nouvelle déstabilisation et le le risque est réel de voir les talibans revenir au pouvoir. C'est ce que nous a confié le fils du commandant Massoud, reçu ce matin par le président Gérard Larcher. Dans le même temps, monsieur le ministre, vous avez rencontré vos homologues de l'OTAN pour aborder le dossier afghan. Parallèlement, des négociations sont en cours entre les États-Unis, la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Inde, le gouvernement afghan et les talibans, négociations dont la France et l'Europe sont exclues. Pourtant, nous serions bien concernés si ce pays sombrait de nouveau dans le chaos. Lorsqu'ils s'exilent, c'est en Europe que vont la majorité des Afghans. En France, les ressortissants de nationalité afghane constituent Abdullah Abdullah, suivant les orientations américaines, négocie avec les talibans au nom du gouvernement afghan. Il nous a confié être personnellement favorable à la participation des Européens aux négociations. Monsieur le secrétaire d'État, la France et l'Europe peuvent-elles intégrer la table des négociations sur le devenir de l'Afghanistan ?

affaires européennes. Monsieur le sénateur Jacques Le Nay, vous avez tout à fait raison, la situation en Afghanistan est extrêmement préoccupante. La décision de retrait des troupes américaines n'est pas remise en cause, mais sa date reste incertaine, alors même qu'approche l'échéance du 1 mai.

devait être conditionné aux progrès de la stabilisation de la situation politique et sécuritaire, et très étroitement coordonné entre alliés. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a également échangé avec la partie afghane pour essayer de débloquer les négociations interafghanes qui ont très peu progressé depuis leur lancement à Doha en septembre 2020. À l'occasion de ces entretiens avec son homologue M. Atmar et avec M. Abdullah Abdullah, qui préside le Haut Conseil pour la réconciliation nationale, le ministre a rappelé le soutien de la France au processus de paix et a insisté pour que les discussions soient élargies et inclusives. Il a souligné qu'il était dans l'intérêt des parties afghanes, notamment des républicains afghans, que l'Union européenne participe

contribuera aussi à cet effort d'élargissement de la participation européenne. La parole comme entre 1996 et 2001. Fawzia Koofi, membre de l'équipe de négociation, a qualifié son pays de « pire pays du monde où naître pour une fille », une déclaration qui en dit long.

Ce soir, l'oracle parlera, mais cet exercice solitaire du pouvoir ne nous fera renoncer ni à notre rôle de parlementaires ni à notre volonté d'associer les Français à la gestion de la crise plutôt que de jouer avec leurs nerfs et de les infantiliser.

étant déjà tendue en temps normal, actuellement on brasse des milliers d'enfants en les répartissant dans d'autres classes, au mépris de la distanciation et des conditions d'enseignement. Nous en sommes là parce que vous avez refusé que les personnels enseignants, en situation de handicap (AESH) et les assistants d'éducation soient vaccinés. Les équipes sont aujourd'hui épuisées, les élus locaux, désemparés, et les familles, inquiètes. Quel est le scénario pour les jours à venir ? Comment la continuité pédagogique sera-t-elle assurée, lorsqu'une classe ou une école, voire davantage seront contraintes de fermer ? des collèges, des lycées et de l'université ? La France va récupérer 2 millions de vaccins dans les prochains jours. doses doivent être destinées prioritairement aux personnels éducatifs, avec un plan précis de vaccination. Les tests salivaires pour les élèves comme pour les personnels doivent s'amplifier et être répétés chaque semaine. Au passage, abandonnez la franchise médicale d'un euro, absolument déplacée dans le contexte. Il faut aussi stopper les suppressions de postes et recruter. À la rentrée 2021, aucune classe ne doit être surchargée.

la sénatrice, dans tout ce que vous avez dit, un point pourrait faire consensus entre nous : c'est une chance pour la France que d'avoir eu ses écoles ouvertes de septembre jusqu'à aujourd'hui. Cela nous singularise dans l'ensemble du monde occidental. En Europe et dans les Amériques, très peu de pays l'ont fait.

la réplique. Monsieur le ministre, j'ai cru un instant ce midi que le Gouvernement allait reconnaître ses erreurs. Il n'en est rien, et j'en suis vraiment navrée. Si vous voulez l'unité nationale, accédez à la demande des enseignants et des personnels éducatifs d'être vaccinés. Si vous voulez l'unité nationale, cessez de fermer des classes à la rentrée. Tout le monde vous le demande, tant dans cet hémicycle que dans le pays. Quand allez-vous enfin l'entendre ?

nationale des étudiants de France (UNEF) a confirmé très tranquillement qu'elle organisait bien des réunions réservées aux personnes de couleur. Lorsque des voix se sont élevées pour dénoncer ces réunions selon la couleur de peau, l'UNEF a persisté et a signé. Non seulement l'UNEF s'obstine, mais des responsables publics n'hésitent pas à justifier une pratique dont on imagine le tollé qu'elle aurait à juste titre suscité si une association ou un syndicat en France avait organisé, à l'inverse, des groupes de parole réservés aux blancs. Bien sûr, les membres du Gouvernement se sont exprimés sur cette dérive. M. Blanquer et Mme Schiappa y sont allés de leur couplet. La condamnation, chaque fois, s'est voulue ferme, dans les propos en tout cas Le Gouvernement ne laissera pas faire », « Tout cela est inacceptable », a-t-on répété à l'envi. Et pourtant, il n'a été question ni d'engager la moindre procédure de poursuite contre une telle pratique qui à l'évidence relève de la loi pénale, ni de suspendre ou de conditionner la subvention que verse l'État à ce syndicat. Pis, nous avons appris dernièrement

comment pouvez-vous afficher une position de fermeté impeccable en façade, et en même temps refuser toute action contre un syndicat qui porte atteinte de manière si claire et si délibérée aux valeurs de notre République ?

et de la participation citoyenne. Monsieur le sénateur Bonhomme, vous interrogez le Gouvernement sur la nomination d'un représentant de l'UNEF au sein du Conseil économique, social et environnemental. de cette nomination, ce que vous remettez en cause, au fond, c'est la réalité de la reconnaissance de la représentativité de l'UNEF. Le Gouvernement- vous l'avez d'ailleurs fort justement rappelé -a eu l'opportunité de s'exprimer par la voix de nombre de ses représentants pour condamner sans la moindre

Le CESE est la chambre de la société civile organisée et de la participation citoyenne. La société civile organisée, présente au CESE, est nécessaire à la vitalité de notre démocratie. Cette nouvelle répartition des sièges

ne le faites pas

mais la réalité est tout autre. Il semble bien que le chiffre que vous citez ne prenne pas en compte toutes les absences liées à la covid, celles-ci augmentant malheureusement tous les jours. En effet, dans bien des établissements du primaire comme du secondaire, des enseignants absents ne sont pas remplacés, et cela désormais sur de longues périodes. Face à cela, les professeurs des écoles organisent au mieux le service, surchargeant parfois les classes pour accueillir des élèves des maîtres absents et provoquant ainsi un brassage favorable à la propagation du virus. Nous pouvons comprendre que la pandémie actuelle complique les conditions de recrutement d'enseignants supplémentaires pour faire face à la situation de plus en plus préoccupante. Mais, monsieur le ministre, le manque chronique d'enseignants remplaçants était déjà connu et ne pouvait qu'être aggravé par la crise sanitaire. Nous l'avions dit lors du vote du budget 2021 : il fallait créer plus de postes pour assurer le remplacement des enseignants dont on pouvait aisément prévoir qu'ils seraient malheureusement frappés eux aussi par la contamination. Puisque la doctrine du Gouvernement est de maintenir les écoles ouvertes coûte que coûte, pourquoi ne pas avoir anticipé des moyens nécessaires lors de la préparation de la rentrée 2020 ? D'ailleurs, nous vous demandons de publier les vrais chiffres du taux de remplacement dans chaque académie, car il semble bien qu'une certaine opacité règne dans ce domaine. Aujourd'hui, la situation est difficile pour les enseignants, et elle se complique considérablement pour les enfants qui, du fait du confinement, ont déjà perdu de nombreuses heures de cours et qui sont de plus en plus nombreux à être en situation de décrochage scolaire. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour pallier dès à présent les absences des enseignants non remplacés ? Comment envisagez-vous la période qui nous sépare de la fin de l'année scolaire ? Enfin, comment préparez-vous la rentrée 2021 dans ce contexte ? La parole

encourent de lourdes sanctions financières, mais elles avaient obtenu un délai. Or en ce début d'année 2021, la banque BNP Paribas, qui s'est vu infliger une amende de plus de 9 milliards de dollars en 2014, menace de façon plutôt énergique de clôturer ces comptes unilatéralement et sous deux mois, y compris quand il y a un prêt immobilier en cours, au prétexte que ces souscripteurs ne peuvent produire ce fameux numéro. En 2018, sur l'initiative de Jacky Deromedi, le Sénat a voté à l'unanimité une résolution invitant le Gouvernement à la mise en oeuvre d'une action diplomatique tendant à obtenir un traitement dérogatoire pour les Américains accidentels leur permettant soit de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite, soit d'être exonérés d'obligations fiscales américaines. Or l'ensemble des services de l'ambassade étant fermés depuis mars 2020 en raison du contexte sanitaire,

Les banques ne peuvent méconnaître cette difficulté insurmontable. Les Pays-Bas ont d'ailleurs abordé le sujet le 16 février dernier, lors de la réunion des ministres européens des finances. Leur ministre s'est alors engagé devant les parlementaires à ouvrir une négociation bilatérale avec son homologue américain. Monsieur le ministre, cette situation et les menaces dont sont victimes nos compatriotes nécessitent une action volontaire auprès de la nouvelle administration Biden, que nous savons attachée au partenariat transatlantique. Pouvez-vous faire le point sur l'avancement de ce dossier, et faire en sorte que le harcèlement de certaines banques cesse ?

depuis 2013, les gouvernements successifs se sont mobilisés, avec d'autres gouvernements européens, pour faire en sorte que ceux que nous appelons les Américains accidentels puissent renoncer plus facilement à la nationalité américaine quand ils le souhaitent. Un guichet spécial a d'ailleurs été mis en place par l'ambassade et le consulat avant la période de covid

pour les résidents fiscaux américains qui ne bénéficient pas du numéro d'identification fiscale, numéro dont vous avez rappelé la difficulté, et parfois l'impossibilité qu'ils avaient à le trouver ou à le retrouver. Ces codes pourront être utilisés dès la campagne de collecte 2021. Par ailleurs, ils permettront de mieux cerner les difficultés liées à la non-obtention des numéros d'identification fiscale nord-américains et de faciliter leur résolution. Je souhaite aussi indiquer que rien ne justifie une fermeture de compte sur le seul fondement qu'un client est américain, qu'il soit ou non américain « accidentel », ou qu'il est dans l'impossibilité de fournir un numéro d'identification fiscale, qui, de plus, est un numéro d'identification fiscale à l'étranger.

Dès le début du premier confinement, les acteurs locaux ont multiplié les initiatives et mobilisé de nombreuses ressources pour protéger leurs concitoyens, maintenir les services publics et soutenir les tissus économique et associatif. Cette crise produit actuellement un choc violent sur les finances des collectivités locales. Ses répercussions dans le temps seront irréversibles. Dans ce contexte, l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur Cette réforme s'applique aux dépenses effectuées dès ce début d'année. Ainsi, pour l'ensemble des bénéficiaires du FCTVA, les dépenses 2021 et au-delà seront traitées dans le cadre de nouvelles modalités de gestion. Du fait de cette réforme, des ajustements ont été opérés. À compter de cette année, les dépenses inscrites sur les comptes 211 et 212, « Terrains » et « Agencements et aménagements de terrains », ainsi que les travaux d'investissement réalisés en régie ne bénéficieront plus de la compensation. À la grande surprise des élus et de leurs associations, l'élaboration, la modification et la révision des documents d'urbanisme ne seront plus éligibles non plus. Ces dépenses substantielles sont souvent amorties sur une durée de dix ans et pèsent de façon importante sur le budget des collectivités. L'incidence de ces pertes d'éligibilité du FCTVA sera extrêmement dommageable pour le bloc communal, qu'elles concernent les documents d'urbanisme indispensables au développement des territoires ou les aménagements de terrains, notamment dédiés au sport. Monsieur le ministre, à la date du 15 avril, les éléments nécessaires à la préparation budgétaire auront-ils été transmis aux collectivités ? Cette date demeurera-t-elle inchangée ? Surtout, quelles mesures entendez-vous prendre pour rétablir l'éligibilité au FCTVA des documents d'urbanisme et des aménagements de terrain ? La parole est à M. le ministre

le ton quelque peu révolté de votre question, dans la mesure où les dépenses liées aux documents d'urbanisme représentent 0,3 % du total du FCTVA. Vous conviendrez donc qu'elles ne constituent pas la majeure partie de cette allocation de 6 milliards d'euros. Nous aurons l'occasion, dans les prochaines semaines et les prochains mois, de travailler sur ces sujets et de perfectionner le

Ils m'ont fait part de leur grande inquiétude, à trois mois du baccalauréat, au sujet de l'épreuve du grand oral. Cette épreuve finale, inédite, est la grande nouveauté du baccalauréat. Elle est déterminante, dotée d'un coefficient important. Les lycéens la travaillent et se montrent studieux, car ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cependant, comment peut-on se préparer à une épreuve dont on ne connaît pas les modalités ? Cette inquiétude est partagée par tous. Les professeurs, formés tardivement, sont écartelés entre la nécessité de terminer le programme et celle de préparer les élèves à l'oral.

De plus, la situation sanitaire impose à certains lycées de fonctionner de manière hybride, en présentiel et en distanciel. Les élèves n'auront donc pas les mêmes conditions de préparation à cet examen, pourtant national, ce rite de passage fort dans la vie d'un jeune adulte.

Cette différence de traitement entre les élèves constitue une rupture d'égalité devant l'examen. Monsieur le ministre, les jeunes, les parents, les professeurs et les élus locaux m'interpellent sur l'urgence de soutenir la jeunesse.

Depuis l'annonce du programme d'accompagnement des « 1 000 premiers jours de l'enfant », nous ne pouvons reprocher à M. Adrien Taquet de manquer d'ambition en matière de petite enfance et de soutien à la parentalité. Cependant, cet intérêt masque mal les difficultés éprouvées sur le terrain, que ce soit par les familles à la recherche de solutions d'accueil pour leur jeune enfant

qui déréglementera les conditions d'accueil des jeunes enfants, en procédant par ordonnances et par décrets. Réduction de l'encadrement,

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a rendu un avis plus que réservé sur ces perspectives. Le rapport du groupe d'experts réunis autour de Boris Cyrulnik préconise un accueil réalisé par des professionnels qualifiés pour garantir le développement et

égard, l'année 2021 sera décisive, comme vous l'avez rappelé. Elle verra, en effet, l'aboutissement de la réforme des règles applicables aux modes d'accueil du jeune enfant, après plus de deux ans de concertation et de travail. Ces nouvelles règles doivent permettre aux professionnels

à part dans la Manche, il a été repéré partout en France. Le loup devient un véritable fléau dans nos campagnes, étendant son territoire à la recherche de nourriture. L'homme ne lui fait plus peur. Dans le Var, à La Verdière, ce sont 300 bêtes du troupeau de l'éleveur local qui ont été tuées en 2020. Le loup est même entré dans la bergerie. Dans le Var, toujours en 2020, ce sont 368 attaques, 1 156 bêtes victimes et 13 meutes qui ont été identifiées. Ces chiffres croissent chaque année. Outre le coût financier, une profonde lassitude pèse sur les éleveurs. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge, faute de se sentir soutenus par les pouvoirs publics. La présence du loup pose également la question de la sécurité alimentaire. Quand le pastoralisme disparaît dans nos territoires, alors que nous prônons le refus des élevages intensifs,

puisqu'il n'a plus de prédateur, hormis l'homme ? Les brigades loup et les louvetiers n'abattent que très peu de bêtes, faute de moyens et d'autorisations. Nous devons non seulement organiser un vrai décompte de la population de ce prédateur, mais aussi ajuster les autorisations préfectorales de tirs de prélèvements et faciliter les tirs de défense pour les éleveurs. Monsieur le ministre, les éleveurs dans nos communes pastorales sont excédés. Montrez-leur que vous les entendez, avant qu'il ne soit trop tard.

Vous verrez des dizaines de bêtes au sol, égorgées, dépecées, à moitié dévorées, parfois encore vivantes et en train d'agoniser. Je ne pense pas que la cause animale et la biodiversité y gagnent beaucoup.

Nous n'avons pas été surpris par les chiffres que le conseil d'administration de France compétences a dévoilés. En effet, au début de l'année 2018, lors de l'examen au Sénat du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avions tenté d'alerter le Gouvernement sur le problème du financement de la formation professionnelle et sur le devenir du 1 % formation. À l'époque, toutefois, votre volonté de recentralisation l'avait emporté, aux dépens du paritarisme et des compétences des régions. Aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes, et les salariés comme les partenaires sociaux sont inquiets. Le manque de financement s'élèverait à près de 5 milliards d'euros pour la période allant de 2020 à 2023, et il pourrait atteindre 10 milliards d'euros sous

Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer comment le Gouvernement compte traiter ce sujet important qu'est le financement de la réforme de la formation professionnelle ? La parole

Par ailleurs, l'augmentation du nombre des contrats d'apprentissage a causé une hausse des dépenses qui sont liées à leur prise en charge. Or nous comptabilisons 500 000 contrats d'apprentissage en 2020, grâce au plan « Un jeune, une au plan « Un jeune, une solution », malgré le contexte de la crise. C'est un record historique. Je rappelle qu'Élisabeth Borne et le Premier ministre

un éventail extrêmement large de formations. Depuis la rentrée, Pôle emploi ou les employeurs peuvent également abonder le CPF pour financer le reste à charge

heures. Mes chers collègues, pour l'organisation du débat qui suivra la déclaration du Gouvernement relative à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre,

les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le délai limite pour les inscriptions de paroles dans le débat pourrait être fixé à demain, onze heures.

Madame la ministre, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste y souscrit totalement. Pour autant, cet article ne mentionne pas seulement le principe de laïcité, mais bien un ensemble de principes que le fonctionnaire doit respecter dans l'exercice de ses fonctions,

et obligations, dont certains ont été précisés et rappelés dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, nous proposons donc d'étendre l'obligation de formation des fonctionnaires, et non de la restreindre au seul principe de laïcité.

Si l'on peut convenir que les exigences minimales de la vie en société, à savoir la construction du vivre ensemble, nécessitent des mesures tendant à renforcer le respect des principes de la République, on ne peut omettre d'inclure parmi ces exigences la reconnaissance et la compréhension des diversités, notamment culturelles et religieuses, qui ont fondé la communauté nationale française. L'article 1 comporte un certain nombre d'avancées, notamment parce qu'il crée une formation au principe de laïcité pour les fonctionnaires et institue un référent laïcité dans les administrations de l'État, les collectivités territoriales

de la religion -et de sa nécessaire mise en perspective avec la laïcité et les valeurs républicaines dans leur ensemble. Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

Ces approches plurielles permettraient de distinguer efficacement ce qui relève du fait religieux dans sa diversité confessionnelle, culturelle et historique, qui est légitime, des tendances « exclusivistes » et séparatistes à prohiber.

si telle est la dénomination retenue par notre Haute Assemblée. Pourquoi faudrait-il une formation spécifique pour ces référents ? Pour deux raisons. La première est que les fonctionnaires seront formés aux principes de laïcité, mais que le référent laïcité pourra ne pas être un fonctionnaire et pourrait donc ne pas avoir bénéficié de cette formation de droit commun. La seconde est que les référents laïcité doivent être mieux et davantage formés que ce que prévoit la formation de droit commun. Le référent laïcité doit bénéficier d'une formation renforcée en comparaison de celle qui est dispensée à l'ensemble des agents. Tel est l'objet de cet amendement de bon sens. nous voulons aborder les questions pratiques, les sujets du quotidien auxquels seront confrontés les référents laïcité.

Être référent est une obligation qui prend du temps. Lorsque l'on est également un agent en activité, il faut pouvoir concilier son activité professionnelle et cette fonction de référent. Pour permettre aux fonctionnaires qui remplissent cette mission de le faire dans les meilleures conditions, nous proposons qu'ils puissent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence. Nous proposons également que les compétences acquises au titre de ces fonctions de référent soient valorisées et prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.

Mme Goulet vient de rappeler l'importance du travail réalisé par cet observatoire : nous avons le sentiment qu'il est aujourd'hui le mieux placé pour répondre aux attentes des référents

dans chaque établissement de santé. En lien avec le référent laïcité de chaque agence régionale de santé, ou ARS, ces deux référents laïcité auront pour mission d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout membre du personnel qui qui le consulte. La mise en place d'un tel dispositif est de nature à faciliter la résolution d'éventuelles questions et problématiques relatives à la mise en oeuvre de la laïcité et de la gestion du fait religieux à l'hôpital. Quel est l'avis de la commission

Christian Redon-Sarrazy. Ce que nous proposons est assez simple. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires garantit la liberté d'opinion aux fonctionnaires. Nous proposons d'y ajouter la liberté de conscience. On nous rétorquera sans doute que la liberté de conscience est garantie à tout citoyen et qu'une telle précision n'est pas nécessaire. Mais la liberté d'opinion est également garantie à tout citoyen ; le législateur a néanmoins souhaité la mentionner explicitement dans le statut général de la fonction publique. Nous proposons cette évolution pour deux raisons. Premièrement, la loi de 1983 interdit de faire des distinctions entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions religieuses ; il serait cohérent d'y inscrire, au préalable de cette interdiction, que la liberté de conscience est garantie aux fonctionnaires. Deuxièmement, par cet ajout, nous souhaitons affirmer clairement que la réaffirmation du principe de laïcité et d'obligation de neutralité ne remet nullement en cause la liberté de conscience. Quel est l'avis de la commission

Autrement dit, derrière la remise en cause de la laïcité, c'est la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité qui est attaquée, car elle représente tout ce qu'ils abhorrent. En guise de réponse à ces attaques, on entend régulièrement qu'il faudrait réaffirmer le principe de laïcité.

Faire vivre la laïcité, c'est évidemment faire appliquer les lois et règlements qui la régissent, mais c'est aussi déployer les outils qui assurent la pédagogie de la laïcité. Tel est le rôle conféré à l'Observatoire de la laïcité

Aussi, cet amendement vise à donner à l'Observatoire une assise législative et, ce faisant, à conforter sa place dans le champ institutionnel, à élargir le périmètre de ses attributions et à renforcer sa composition.

Commission consultative nationale des droits de l'homme ou encore la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Ainsi, nous entendons souligner la singularité de l'acceptation française du principe de laïcité.

cette valeur ! Vous contestez l'initiative que nous prenons, faute de proposition du Gouvernement

aux préfets une circulaire relative à la lutte contre les dérives sectaires, reprenant ces éléments et leur demandant la plus grande vigilance, en écho au rapport que m'ont remis la police nationale, la gendarmerie nationale et la Miviludes il y a de cela deux semaines.

des sujets dont vous avez discuté hier et dont nous allons continuer de débattre : la systématisation de ces référents, l'animation du réseau qu'ils constituent, ou encore le caractère obligatoire de la formation à la laïcité

d'éclairer le Gouvernement et, peut-être, de coordonner l'ensemble des structures existantes, comme celles qui ont été mentionnées précédemment. Bien entendu, les parlementaires y seraient le cas échéant associés. Ce sont là des pistes de travail et de réflexion et, comme je l'ai indiqué, le Premier ministre fera connaître son arbitrage dans les prochaines semaines.

commis « contre » les agents hospitaliers, mais bien « par » les agents hospitaliers. Il amène les référents laïcité qui exercent dans les hôpitaux à avoir l'obligation d'alerter l'agence régionale de santé, l'ARS, sur tout manquement au principe de laïcité commis par un agent public hospitalier. On se retrouve donc avec un article 1 qui jette la suspicion sur les agents de la fonction publique hospitalière, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les personnels administratifs, en laissant entendre qu'ils transgresseraient le principe de laïcité plus que tous les autres agents publics. En conséquence, il faudrait les soumettre à un régime spécifique d'alerte auprès des agences régionales de santé. Pour ce qu'il insinue à l'égard de l'ensemble de ces personnels, en particulier dans la période que nous connaissons et au regard de ce que nous leur devons, cet article nous semble totalement choquant et nous en demandons la suppression. Par ailleurs, cet article procède à une confusion sur le rôle du référent laïcité. Nous l'avons dit depuis un certain a une mission de conseil auprès des agents. Lui imposer, comme le prévoit l'article, une obligation de signalement en cas de manquement aura un effet contre-productif, puisque cela pourrait tout simplement décourager les agents de venir requérir ses conseils. C'est au chef de service d'intervenir en cas de manquement au principe de laïcité- cela peut arriver -, en mettant en mouvement le régime disciplinaire applicable à l'agent. Ce n'est pas au référent laïcité, auquel l'agent doit garder toute confiance, de le faire.

Cette proposition de supprimer l'obligation, pour les référents laïcité des établissements de santé, d'alerter l'ARS de tout manquement dans un délai de quinze jours est motivée par la volonté de préserver l'équilibre de l'article 1 et de ne pas créer au sein de la loi de confusion sur le rôle de référent laïcité. Toutefois, puisque la rédaction ne nous apparaissait pas satisfaisante pour les raisons mentionnées, nous proposons par ailleurs un amendement de repli, qui nous semble pouvoir constituer un compromis, afin de renforcer la connaissance des manquements à l'exigence de neutralité, ainsi que le traitement des situations visées. Cet amendement de repli a pour objet de conserver dans le projet de loi un article relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements de santé et les ARS sur les manquements à l'exigence de neutralité des agents publics.

les agents référents laïcité dans les hôpitaux auront toujours comme mission de signaler aux ARS les manquements de leurs collègues. C'est donc un contresens par rapport au principe même de référent laïcité, qui est là pour conseiller l'agent, pour apporter un éclairage, et non

à l'exigence de neutralité des agents publics. Au regard des difficultés auxquelles sont confrontés les établissements de santé, la compétence première est bien celle du directeur d'établissement, même si l'ARS pourra exercer un suivi rapproché.

publics.

ainsi préférable que la suspension de l'acte soit décidée par un juge, dans le cadre d'une procédure d'urgence justifiée par l'importance des principes auxquels il est porté atteinte, plutôt que par le préfet.

Un tel dispositif est évidemment souhaitable, mais il soulève une interrogation quant à la rédaction retenue. En effet, comment distinguer une atteinte d'une atteinte grave à la neutralité des services publics ? Peut-on envisager qu'une atteinte à ce principe si fondamental ne soit pas grave par nature ? Toute atteinte à ce principe doit être considérée comme inacceptable. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer la qualification « gravement » pour ce qui concerne l'atteinte portée au principe de neutralité des services publics.

Il prend racine à Strasbourg, grâce à la complaisance et à la complicité des élus municipaux islamo-gauchistes. Ainsi, 2 500 000 euros ont été versés par la municipalité pour la construction d'une mosquée géante- il s'agit de la plus grande d'Europe -, à une association extrémiste turque, Millî Görüs. C'est exact ! Cette association, toujours pas dissoute, a refusé de signer votre charte de l'islam, madame Schiappa. Elle n'a manifestement pas la reconnaissance du ventre elle aurait pu la signer pour remercier votre ministère de lui avoir accordé une subvention de 2 500 euros au titre de la politique de la ville et de 22 400 euros au titre de la prévention de la délinquance ... Entre vos subventions à une association islamiste et la nomination,

votre capitale européenne ! Il est loin le temps où le général Leclerc libérait la ville de l'envahisseur en dressant le drapeau français sur sa cathédrale. Un contrôle de légalité du préfet s'impose sur une telle décision de la municipalité strasbourgeoise. Tout y est : l'ingérence étrangère, l'expansionnisme islamiste et la collusion généralisée de la classe politique Le mécanisme de veto ou de substitution par l'autorité préfectorale va dans le bon sens. Néanmoins, il faudra régler, au moment des lois de finances, le problème des diminutions des moyens en personnel dans les préfectures pour ces contrôles qui tardent et sont moins précis. Le plan Préfectures nouvelle génération portait des promesses sur ce point, mais leur réalisation n'est toujours pas au goût du jour. C'est pour une meilleure effectivité de la loi que je propose de retirer le terme « gravement » de cet article. En effet, avant d'arriver au stade de la mosquée géante, l'islamisme a progressivement grappillé du terrain et s'est installé à Strasbourg, comme ailleurs, grâce à de nombreuses décisions non sanctionnées par le tribunal administratif. Dans le respect de la libre administration des communes, et avec le respect qui est dû aux élus locaux, dont je fais partie, il faut donner à l'État les armes de la reconquête sans sourciller dans les termes. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Le projet de loi répond qu'il s'agit des actes portant gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics. Il nous semble que le terme « gravement » est impropre à cet effet, mais pas pour les raisons évoquées par nos collègues. Le débat n'est pas de distinguer les atteintes qui sont graves et celles qui le seraient moins ; il ne s'agit donc pas de dire qu'il y aurait des atteintes au principe de laïcité qui seraient acceptables. Le déféré « accéléré » est une procédure qui ne préjuge pas de la décision sur le fond. C'est au moment de la décision sur le fond que le juge administratif appréciera de la gravité de l'atteinte. Au stade de la suspension, la question est de savoir si l'atteinte est manifeste ou non. Si elle l'est, il y a déféré « accéléré » ; si elle ne l'est pas, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous proposons de remplacer le terme « gravement » par « manifestement

de ce qui est en cause est moins important que le fait de préciser « gravement ». Le caractère plus ou moins manifeste de l'illégalité ne semble donc pas de nature à justifier un recours à une procédure juridictionnelle accélérée.

ont donné à certains de leurs élus une délégation de fonction pour exercer différentes attributions relatives aux cultes, à la spiritualité ou aux religions- il y avait tout un vocabulaire dont je vous passe l'ampleur. J'ai écrit à M. le ministre de l'intérieur et j'ai déposé une question écrite- la question n° 17 302 du 16 juillet 2020 -en lui demandant d'exercer sur les préfets une aimable

il n'y a que l'État qui a la possibilité de faire respecter les articles de la loi de 1905 relatifs à la police des cultes. Les collectivités n'ont aucune compétence dans ce domaine et n'ont aucune raison d'avoir des élus délégués aux

des cultes. Et vous me dites que l'on pourrait passer outre et qu'il s'agit de la liberté du préfet. Je ne comprends donc pas la cohérence de votre propos. Je crois que si l'on tient vraiment à ce que les principes de la République soient défendus, il faut donner une mission spécifique aux préfets pour le contrôle des actes des collectivités. J'ai réussi à trouver une place pour cette décision dans le code général des collectivités territoriales

M. Didier Marie. Nous proposons, par cet amendement, de compléter la charte de l'élu local qui figure dans le code général des collectivités territoriales, pour y inscrire noir sur blanc le principe de laïcité et l'interdiction pour tout élu local, à ce titre, de manifester ses opinions religieuses dans l'exercice de ses fonctions. L'Assemblée nationale a utilement précisé les choses concernant les conseillers municipaux exerçant par délégation des fonctions d'officier d'état civil, mais il y a lieu d'aller plus loin et de prévoir que tout élu local doit être soumis au respect du principe de laïcité lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. Qu'il siège dans un conseil d'école ou qu'il s'exprime lors d'une remise de prix d'une compétition sportive, l'élu y représente la collectivité. À ce titre, il ne peut manifester ses opinions religieuses et le principe de laïcité doit s'appliquer, quel que soit son mandat- municipal, départemental ou régional -, son rang ou sa délégation. Je précise, pour éviter toute mauvaise interprétation, que serait seul mentionné dans la Charte de l'élu local le principe de laïcité. Il n'y a pas lieu d'appliquer aux élus locaux l'obligation de neutralité,

municipaux et des commissions permanentes du département ou de la région. Ainsi, il vise à étendre les dispositions de l'article 2 , afin d'inscrire dans la charte de l'élu local la nécessité, pour l'élu local, de ne pas porter de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse durant les réunions des organes délibérants des collectivités. Pourquoi s'agit-il d'un amendement de cohérence ? Parce que la réglementation de nos assemblées nationales, qu'il s'agisse

quelconque opinion : est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique.

Cette exigence républicaine héritée de l'histoire parlementaire contribue à assurer la sérénité requise lors des délibérations du Sénat. » Mes chers collègues, demander, dans notre République laïque, un minimum

à titre tout à fait personnel, je suis favorable

dans l'ensemble de leur vie publique. Bien entendu, les conséquences de son adoption seraient considérables. Nous souhaitons pouvoir continuer à fêter la Saint-Michel des parachutistes, la Sainte-Geneviève des gendarmes ou la Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers

à l'encontre des grands principes que nous trouvons au faîte de nos grands textes, comme d'ailleurs dans les différents règlements intérieurs de nos assemblées parlementaires et des collectivités locales ? Monsieur Paccaud,

ce qui est, à mon avis, contraire à la loi, devrait s'habiller en civil pour rencontrer, dans le cadre de sa délégation, un homme d'Église, quel qu'il soit.

nous aurions préféré que la loi de 1905 soit appliquée dans toute sa rigueur et que le préfet défère systématiquement devant les tribunaux administratifs les actes des collectivités qui ne sont pas conformes à l'esprit de la République. La parole est

J'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne s'agit pas, avec notre amendement, de décréter que tous les élus doivent faire preuve de neutralité. On leur demande de respecter les principes de laïcité, ce qui signifie que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'ont pas à faire valoir leurs convictions religieuses. Cela ne les empêchera pas, cher Loïc Hervé, de citer tel philosophe, tel écrivain ou telle référence.

l'habit ne fait pas le moine, des moines peuvent être élus dans nos conseils municipaux. Pour autant, ils peuvent tout à fait respecter le principe de laïcité en ne faisant pas valoir leurs convictions religieuses

on peut tout à fait exprimer ses idées, quelles qu'elles soient, sans porter de vêtement militant.

ne sont plus l'incarnation des choix politiques et de la démocratie. C'est en cela que les dispositions de ces deux amendements

Je rejoins les propos de mes deux collègues Bas et Brisson : cette liberté ne doit pas être restreinte, ni dans le champ religieux ni dans le champ politique. Elle doit être la plus large possible.

Cet article a été voté en souvenir de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, par laquelle la République s'est sabordée à Vichy, et j'honore la mémoire des quatre-vingts parlementaires qui se sont S'il y a quelque chose de fondamental dans notre démocratie, dans la République, c'est que l'on peut y discuter de tout, sauf de la forme républicaine du Gouvernement. Les partis politiques peuvent se constituer librement, sans aucune entrave.

l'abrogation de la loi de séparation des Églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État pour l'instauration du règne social du Christ Roi ». Tel est l'objet de ce parti politique, que vous financez, mes chers collègues

par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. Le contenu de la propagande électorale ne peut pas faire l'objet d'un contrôle par l'administration, sauf à ouvrir la voie

comporte une mention qui serait de nature à contrevenir aux principes de laïcité ou de souveraineté nationale. Or le contrôle du préfet, lors de la prise de candidature, est formel : son rôle consiste non pas

par les candidats, de principes républicains, afin de priver des candidats dits « communautaires » de financement. S'il est possible d'imaginer une conditionnalité du remboursement et de la propagande qui pourrait être pertinente, celle-ci devrait se fonder sur des critères objectifs et rationnels, avec des définitions recueillant l'assentiment et le consensus

nos concitoyens contre l'émergence de listes communautaristes. Bien évidemment, une liste remettant en cause la forme républicaine du Gouvernement aura toujours le droit de se présenter : les monarchistes, par exemple, ont toujours le droit d'être candidats à l'élection présidentielle. Pour autant,

en expliquant qu'elle était majeure. Mais pourquoi, depuis le 8 novembre 2019, n'avez-vous pas proposé qu'elle soit discutée ici ? Ce premier point m'intrigue.

qui semble être, selon un certain nombre de spécialistes, une officine de l'AKP, avait présenté aux cantonales, dans le Bas-Rhin, des candidats. Il en a ensuite présenté, en 2017, dans plus de cinquante circonscriptions. Pourquoi ? Tout simplement pour bénéficier des financements publics

listes de ce parti se sont présentées, en France, à ces élections législatives. Elles ont accédé au financement public,

à ces pays étrangers, qui veulent saper l'unité républicaine et qui font preuve d'un entrisme politique incroyable dans une démocratie comme la nôtre, qu'ils n'ont pas leur place dans notre République.

et trouver des solutions pour se prémunir de leur présence lors des élections.

les idées qu'elles véhiculent. Je crois que l'on combat mieux le séparatisme par l'action et le débat politique, y compris en menant ces débats au moment des élections.

que celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

45. Bientôt le débat sur cet article sera plus long que celui qui porte sur les amendements eux-mêmes ! Par conséquent, mes chers collègues, il faut en revenir à une lecture sage de la Constitution.

que l'on en tire les conséquences à l'avenir.

les censures du Conseil constitutionnel, on ne fera plus rien du tout. Comme disait le général de Gaulle, en France, la seule Cour suprême, c'est le peuple français.